La séance est reprise. La parole est à madame Marie-Pierre Richer pour une mise au point, au sujet d'un vote. Merci, monsieur le Président, je souhaite faire la mise au point suivante sur le le scrutin public numéro 270. Ma collègue Elsa chaque souhaitait s'abstenir. À été donné de votre mise au point, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans la liste politique du scrutin. L'ordre du jour appelle le débat sur la pollution lumineuse, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. La parole et tout d'abord à l'orateur de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui a devancé ce débat. Madame Annick Jacquemet au nom de cet office pour huit minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre Mesdames et messieurs les sénateurs. Le 26 janvier dernier, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a adopté la note scientifiques sur la pollution lumineuse dont il m'avait chargé et a souhaité que ce sujet fasse l'objet d'un débat public en effet la pollution lumineuse est un phénomène massif en pleine extension au niveau mondial et qui contribue au même titre que d'autres pressions anthropiques au déclin de la biodiversité en outre la pollution lumineuse soulève de réelles préoccupations en matière de santé publique. Je vous renvoie à la note qui en détaille les caractéristiques ainsi que des effets. Face à ce constat, seule une mobilisation collective, à la fois des pouvoirs publics, État et collectivités territoriales. Et des acteurs privés permettra de lutter contre elle. La France a développé une réglementation particulièrement ambitieuse pour limiter les nuisances lumineuses la temporalité de très nombreux éclairage est encadrée et limitée, qu'il s'agisse des éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel des parcs et des jardins des chantiers extérieurs des parkings desservant une activité économique des lumières éclairant le Patrimoine, des éclairages de vitrines de magasins ou encore des publicités et enseignes lumineuses. Par ailleurs la réglementation fixe les prescriptions techniques qui visent à ne pas éclairer le ciel à limiter l'éblouissement latéral à réduire les températures de couleur. Toutefois plusieurs obstacles affaiblissent l'efficacité de ces mesures. D'abord l'application de la législation restent limitées tant que tous les arrêtés ne sont pas pris. celui fixant les seuils maximaux de l'imminence des enseignes et des publicités lumineuses n'a toujours pas été publiés dans l'attente d'un arbitrage ministériel. Je souhaiterais donc savoir Madame la Ministre quand cet arrêté sera publié et quelle version sera retenu puisque selon mes informations de versions avec des ambitions différentes vous ont été proposés. J'ai également constaté que la réglementation actuelle reste incomplète. Ainsi les événements extérieurs et les équipements sportifs font partie du Champ d'application de l'arrêté du 27 décembre 2018. Mais ils ne font l'objet d'aucune prescription de pour de temporalité ni de prescriptions techniques. Autres trous dans la raquette, les exigences en matière de lumière émise vers le ciel ne concerne que l'éclairage de voiries et les parcs de stationnement, alors même que l'éclairage privées représentent souvent une part importante des lumières émises à cet égard un réel travail d'information des consommateurs est amené les fabricants d'ampoules et de luminaires mais également les enseignes de bricolage devrait s'assurer de l'innocuité des sources lumineuses qu'ils vendent et conseiller les consommateurs dans le sens d'une plus grande sobriété lumineuse qui ne se limite pas à la sobriété énergétique. En effet, si les leds ont un rendement lumineux très important et permettent de réaliser des économies d'énergie, leur faible consommation peut devenir un argument pour multiplier les points lumineux alors que leur efficacité énergétique est inversement proportionnel à leur impact sur la biodiversité en raison de leur forte proportion de bleu. Par ailleurs, si des sanctions sont prévues en cas de non respect de la réglementation visant à lutter contre la pollution lumineuse dans les fêtes, elles ne sont jamais appliquées. Une étude récente de la Direction interministérielle de la fonction publique a cherché à comprendre pourquoi la réglementation sur l'extinction nocturne des commerces étaient peu impliqué, alors même qu'elle date de 2013. Cette étude fait les constats suivants, d'abord les maires connaissent mal la réglementation ensuite le contrôle de l'extinction nocturne et fastidieux puisqu'il exige la mobilisation des services municipaux entre une heure et 7h du matin. Il s'agirait donc de sensibiliser les mairies sur la réglementation et leur rôle à travers un support d'information simple et facilement accessibles. De fournir aux collectivités des outils pour communiquer avec les commerçants, tels que des guides pratiques et des courriers type de mettre en avant les bénéfices réputationnel à agir dans la mesure où les Français sont très majoritairement favorables à l'extinction nocturne des commerces en un mot il faut simplifier la tâche des maires qui croule déjà sous les obligations. En ce qui concerne l'action en direction des commerçants. Il convient de leur rappeler la réglementation et les sanctions en cas de non respect et de les sensibiliser à des moments clés comme la création de nouveaux magasins ou encore l'lors de demande d'aide. Par ailleurs, il me paraît indispensable d'associer les fédérations de commerçants pour diffuser l'information sur la réglementation. Le syndicat de l'éclairage doit également se mobiliser pour rappeler les règles d'extinction aux professionnels de l'éclairage les sensibiliser à mettre en place des solutions faciles permettant de gérer l'extinction des vitrines mais également de tous les points lumineux dans les magasins qu'il s'agisse des présentoirs ou encore des enseignes lumineuses. À l'intérieur des vitrines dans le développement et malheureusement en pleine explosion. Au niveau local de nombreuses collectivités ne disposent pas toujours des outils juridiques nécessaires garantissant la pérennité de leur action dans la lutte contre la pollution lumineuse. Je voudrais citer 2 exemples, un nombre croissant de communes éteigne l'éclairage des voiries au coeur de la nuit. Pourtant la responsabilité du maire peut être engagée en cas d'accident. Madame la Ministre, que proposez-vous pour protéger les maires. De même, de nombreuses communes mettent en place des trams noirs qui à l'image des trames vertes et bleues vise à recréer une continuité nocturne pour préserver la faune et la flore qui ont besoin de la nuit. Pourtant de nombreux responsables municipaux ont estimé que le cadre réglementaire de ces trams noir reste précaire, faute de leur mention dans le code de l'environnement. Madame la Ministre partagez-vous cette analyse comment rendre opposable les trams noirs dans des documents d'urbanisme. Si la rénovation des éclairages publics permet de supprimer des installations particulièrement énergivores. Elle ne permet de lutter efficacement contre la pollution lumineuse que si elle s'accompagne d'une réflexion préalable avec les usagers sur la finalité des éclairages et sur leur réelle utilité au regard des besoins avérés des habitants. Il s'agit donc de changer de paradigme en passant d'un éclairage systématique à une adaptation fine, selon le contexte. La pollution lumineuse a également des effets délétères sur la santé humaine qu'il convient de combattre. D'abord, certaines sources lumineuses sont photo toxique dans la mesure où elles échappent à la réglementation qui impose que seuls les lampes du groupe photobiologique égal à 0, c'est-à-dire sans risque ou un risque faible sont autorisés. Il s'agit notamment des lampes torches et des phares de voitures. Par ailleurs, les valeurs limites d'Exposition définies au niveau international date de 2013 et ne prennent pas en compte la sensibilité particulière des enfants et des jeunes adultes. Le 4ème Plan national Santé environnement prévoit l'interdiction par la France des l'aide de groupes à risque supérieur à 1 dans les articles à destination des enfants et dans les lampes frontales. Il précise également que la France portera au niveau européen une demande d'interdiction des phares automobiles à l'aide de groupes à risque supérieur à 1. Madame la Ministre où en êtes-vous dans ses initiatives. Enfin pour terminer, je voudrais insister sur les dangers de dérégulation du cycle circadien liés à l'Exposition à la lumière artificielle bleu dégagé par les éclairage et les écrans en soirée et la nuit et sur la nécessité de mener régulièrement des campagnes de sensibilisation en direction de toute la population et en particulier des enfants et des adolescents. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le. Le président, madame la rapporteure mesdames et messieurs les les sénateurs. 50%. C'est le pourcentage d'augmentation de points lumineux en France en 30 ans. Or nous savons et les études le prouvent la pollution lumineuse, a un impact négatif sur la biodiversité. Elle est aussi devenue un enjeu de santé publique de sobriété énergétique et même de paysages nocturnes de plus en plus de citoyens étant privé de l'observation d'un ciel étoilé. Alors merci, merci madame la rapporteure et les membres de l'Opecst pour votre travail étayée sur ce sujet stratégique, et merci d'ouvrir ce débat aujourd'hui. Ce rapport suit directement le travail réalisé en 2021 sur le déclin des insectes problématique centrale dans la protection de la biodiversité. Mais les enjeux dépassent de loin la simple question des insectes environ un tiers des vertébrés et 2 tiers des invertébrés sont nocturne et dépendent directement de la nuit. Pour les espèces dis urnes comme l'être humain. La nuit est synonyme de repos et est essentiel pour la bonne santé pour les espèces nocturnes les nuisances lumineuses sont une menace directe sur leur activité. Le développement humain, urbain, pardon de ces dernières décennies a entraîné un recours quasi systématique à l'éclairage artificiel. À l'origine d'une pollution lumineuse inédite. La lumière artificielle, nuit à la physiologie et au métabolisme des espèces, ce qui perturbe leur bon développement. Cette pollution a aussi des effets encore plus Direct et observables sur certaines espèces, à savoir la fragmentation de leur habitat. Par exemple une route éclairée peut constituer une véritable barrière hein Francis infranchissable pour des amphibiens aux migrations et à l'inverse les papillons de nuit vont être attirés par l'éclairage et tourner indéfiniment autour jusqu'à épuisement. Sans parler de nombreuses espèces notamment d'oiseaux et d'insectes qui se servent du ciel étoilé pour se repérer et se déplacer. On comprend donc très facilement que l'ampleur de cette pollution est grande. Elle a trop d'impact négatif sur la biodiversité. Elle est source de trop de gaspillage d'énergie et elle est par ailleurs source de gaspillage de beaucoup d'argent. Bien sûr l'éclairage de l'espace public est nécessaire, nécessaire pour se déplacer nécessaire aussi pour certaines activités économiques. Cependant les développements technologiques et les attentes citoyennes en la matière, doivent nous permettre de concilier biodiversité et aussi Cadre de vie. Ce sujet doit devenir une priorité et nous devons l'intégrer à notre manière de penser la ville. L'objectif n'est pas de décroître. Mais d'éviter tout surplus inutile. Certains élus locaux sont précurseurs et ont déjà évolué sur ce sujet, c'est avant tout par souci d'économie budgétaires que les communes en sont venus à réduire leur éclairage. Désormais nos concitoyens soutiennent aussi c'est stratégique pour d'autres raisons notamment des raisons environnementales. En formule en ce sens de nombreuses propositions que j'ai étudié évidemment avec beaucoup d'intérêt. Je souhaite que nous avancions ensemble sur ce sujet et j'ai moi-même des propositions à vous faire. D'abord concernant la publicité lumineuse. La réglementation existe. Nous avons déjà commencé à agir. Puisqu'en octobre dernier, nous avons renforcé la réglementation avec l'obligation d'extinction nocturne sur tout le territoire alors que jusqu'ici, seuls les plus grandes agglomérations étaient concernés. Maintenant il y a la question de l'application de cette mesure et je vous confirme qu'elle n'est pas suffisamment appliqué. Pourquoi. Parce que le système de sanctions nécessite de passer par un juge. Ce qui le rend inopérants, et qui ne pousse pas les maires Je vous propose que nous facilite édition ce contrôle en rendant possible la forfaitisation d'une amende. Ensuite, pour ceux qui ne relève pas de la publicité mais de l'éclairage intérieur et extérieur non résidentiels. La réglementation mérite aussi d'être renforcé. Actuellement, l'éclairage des bâtiments non résidentiels doit être éteint de une heure à 7h du matin je souhaite aller plus loin et fixé l'extinction pour ces bâtiments par exemple une heure après la fin de l'activité et jusqu'à une heure avant la reprise de l'activité. Enfin s'agissant des espaces naturels protégés. J'ai demandé à l'OFB de cibler les contrôles dans les espaces les plus sensibles. Nous pouvons aller plus loin dans la création de tram noir. Aujourd'hui, seuls 15% de notre territoire est indemne de toute pollution lumineuse. Nous devons faire mieux notamment en généralisant les trams noirs dans les espaces protégés. Cela sera intégrée dans la stratégie nationale biodiversité annoncer prochainement. Les opérateurs de transport ont également leur rôle à jouer. Je tiens à ce titre, a souligné la signature d'une charte le 27 mars dernier qu'il conduit à mieux réguler la publicité lumineuse dans les gares les stations et les aéroports, dans le cadre des plans de sobriété des secteurs concernés porté par Agnès Pannier-Runacher et Clément Beaune avec cette charte les opérateurs s'engagent à éteindre 100% de leurs panneaux lumineux dès la fermeture des gares, des aéroports et des métros. D'ici le 1er janvier 2024. Il s'engage également à établir une stratégie de sobriété, de la gestion de leur parc de panneaux lumineux. La RATP s'est engagée à réduire de 35% sa consommation électrique d'ici 2026 la SNCF de 45% d'ici 2031 et ADP de 50% d'ici 2030. Ça, c'est concret, c'est réaliste et c'est efficace. Je suis maintenant prêt à échanger avec vous. À imaginer ensemble de nouvelles mesures capables de faire évoluer notre société vers plus de sobriété lumineuse. Ceci étant Ceci autant pour réduire notre consommation électrique que pour mieux protéger une divorcée une biodiversité de plus en plus menacées. Cela nécessitera une nouvelle fois un travail collectif avec vous parlementaires ainsi que les collectivités locales et tous les acteurs économiques concernés. Car la protection du vivant est une mission qui nous concerne tous, chacun à notre niveau, je vous remercie. Merci madame le Ministre. dans le débat interactif. Chaque orateur. Disposera de 2 minutes, y compris la réplique et avec une possibilité de réponse du gouvernement pour une durée équivalente. Puis possibilité pour le gouvernement de répondre à une réplique pendant une minute et pour l'auteur de la question de répondre à nouveau pendant une minute. Voilà. Nous commençons par madame Annick Billon de l'Union centriste pour 2 minutes. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre madame la rapporteure. Le nombre de panneaux d'affichage traditionnel rétro-éclairé augmente dans le domaine public à Paris par exemple, il est fait état de 1700 panneaux d'affichage. Ces affiches qui fonctionne généralement avec des néons alimenté par un petit moteur branchées sur l'éclairage public ne sont pas moins polluante que les panneaux numériques à technologie LED. De plus en plus de villes, les grandes villes françaises, telles que Colmar, Rouen, Nice et Paris interdisent complètement le déploiement d'écran numérique dans le domaine privé, aussi bien en coeur de ville qu'en périphérie. Ces interdictions sont justifiées au titre de la pollution visuelle et environnementale. Mais en parallèle, la mairie de Paris par exemple installe 180 panneaux numériques dans l'espace public et cela au titre de la sobriété énergétique. Le SNPL Syndicat national des professionnels du numérique s'apprête à déposer une plainte contre la France auprès de la Commission européenne pour entrave à la liberté du commerce et de l'industrie. La jurisprudence et le droit européen reconnaissent l'application du principe de proportionnalité dans le cadre de la réglementation de la publicité extérieure or mobilier urbain mais ce principe de proportionnalité n'est pas appliquée en France. Madame la Ministre, quelle est la position du gouvernement, le ministère de la transition écologique entend-il dans le cadre d'une modification par décret imposé aux règlements locaux de publicité le respect du principe de proportionnalité, comme cela se fait chez grand nombre de nos voisins européens. Je vous remercie. Merci monsieur le le président, mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Billon. Le règlement national prévoit que dans les agglomérations, la publicité est admise mais doit toutefois satisfaire certains critères notamment en matière d'emplacements de densité de surface de hauteur d'entretien et pour la publicité lumineuse d'économie d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses, lesquels sont précisées justement par voie réglementaire. Le règlement local de de publicité permet de définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions minimales du règlement national sous ce principe le règlement local de publicité permet aux collectivités territoriales d'adapter la réglementation nationale en matière de publicité extérieure au regard des enjeux locaux et à la réalité des territoires. Il s'agit ainsi de trouver un équilibre entre des dispositifs ambitieux de préservation des paysages et du cadre de vie et des objectifs de développement économique des territoires. Le principe de proportionnalité et donc naturellement un fondement de l'élaboration d'un règlement local de publicité dans la recherche de cet équilibre sans qu'il soit besoin de l'ériger en principe plus généralement tout encadrement par les collectivités par voie réglementaire d'une activité économique fait l'objet justement d'un examen par les services de l'État dans le cadre du contrôle de légalité et peut faire l'objet D'un contrôle par les juridictions administratives afin que soit vérifiée justement les équilibres entre les différents intérêts, protégés. En l'espèce, la qualité du paysage ou encore du Cadre de vie versus l'activité économique.

les services de l'État travaillent ensemble, je voudrais juste rappeler que dans un rapport publié en 2021, le RT estime que la réduction de l'utilisation des écrans publicitaires lumineux sur une année somme toute normal hors crise sanitaire et guerre en Ukraine. Influerait sur à peine 0,1% du total de la consommation énergétique en France. Donc si le normal d'encadrer l'implantation et le fonctionnement des panneaux numériques ce que ce pourquoi nous sommes tous d'accord, il convient de le faire de manière pragmatique, c'est ce que vous avez voulu. Répondre. À l'instant donc je vous remercie pour cette réponse Monsieur le président, madame la secrétaire d'État mais madame la sénatrice Annick chaque mes, mes chers collègues. Dans un premier temps, je tiens à remercier l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour la programmation de ce débat, oh combien important aujourd'hui. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom du groupe RDSE. En tant que sénatrice et conseillère départementale de la Lozère territoire précurseur en matière de lutte contre la pollution lumineuse puisque le 13 août 2018, le parc national des Cévennes a obtenu de la belle réserve internationale de ciel étoilé, devenant la plus vaste d'Europe. Veeva moi même au coeur de la zone centrale de la réserve ou la noirceur naturel et préserver au maximum je peux témoigner du bien-être que cela procure de pouvoir observer un ciel étoilé Net est-ce un gène extérieur. Qui plus est lorsque l'on connaît les impacts positifs que cela peut engendrer sur la faune, la flore, la santé humaine et la baisse des dépenses énergétiques pour les petites communes. Il me semble à ce propos qu'il est primordial de saluer le travail conséquent réalisés par les acteurs impliqués comme les établissements publics, les syndicats d'électricité et surtout les collectivités locales qui sont à gestion directe. Mon interrogation porte sur le calendrier de mise en vigueur des dispositions indiqué dans l'arrêt du 27 décembre 2018 relatif à la limitation des nus, des nuisances lumineuses. En effet les mise en conformité des installations. Elle dit existantes s'échelonner jusqu'au 1er janvier 2025 avec des échéances intermédiaires. Comme évoqué ci-avant bon nombre de communes se sont engagés très tôt dans une démarche vertueuse pour une réduction drastique de la pollution lumineuse. Ainsi, madame la secrétaire d'État. Avez-vous imaginé un système de bonus incitatifs qui permettrait aux petites communes précurseur d'obtenir un accompagnement technique et financier complémentaire. Par ailleurs, avez-vous mesuré les besoins en ingénierie des communes qui ne sont pas dans des périmètres de parcs naturel et qui peut qui qui peuvent être en difficulté face à l'implication de cet arrêté. Je vous remercie. Merci monsieur le le président, mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Pentel moi je dire je vous remercie de prendre l'exemple des actions qui ont été mises en place dans le parc national des Cévennes que vous connaissez bien et parce que c'est un très bel exemple justement d'initiatives qui pourraient se dupliquer dans d'autres espaces protégés. Vous avez raison, il faut que les collectivités soient incités financièrement à mener des plans ambitieux de lutte contre la la pollution lumineuse. À défaut d'incitation, le risque serait que des, que ces actions restent au stade seulement d'initiative sans connaître généralisation alors que c'est bien par cette mise à l'échelle que nous réduirons réellement l'impact de la pollution lumineuse sur la consommation d'énergie et la biodiversité des efforts ils doivent être récompensés en réalité aujourd'hui nous avons un double bonus déjà pourquoi. L'économie d'énergie recherché par les élus locaux quand ils rénovent leur part d'éclairage et aussi une économie financière sur la facture, on voit bien que le signal prix apporte un réel effet levier et je partage l'avis de Madame Billon c'est pas tant pour la baisse d'énergie généré les subventions obtenues dans le cadre du Fonds Vert ensuite l'incitation financière, c'est tout l'objectif justement du Fonds Vert que nous avons officiellement lancé en janvier dernier qui connaît un réel succès. Il permet de financer 40% d'un projet et ainsi de déclencher des investissements de la part des collectivités qui ne se serait peut être pas. Sans cet accompagnement et cet investissement leur permettra de réaliser des économies d'énergie et donc des économies aussi financière. C'est un cercle vertueux pour les collectivités. J'aurais d'ailleurs l'occasion de vous présenter un bilan du Fonds Vert plus détaillée je pense un peu plus tard parce que je pense qu'il y a des questions qui reviendront sur le sujet. Merci Madame le Ministre. La parole est à monsieur Jean-Claude Lenglart pour les républicains pour 2 minutes. Merci monsieur le président, madame la ministre madame le rapporteur, mes chers collègues. L'émergence du problème public de la pollution lumineuse date de plus de 50 ans. La prise de conscience des enjeux de la pollution lumineuse et de ses nombreuses aux conséquences néfastes et variées a toutefois été accélérée par l'augmentation du prix de l'énergie. En quelques mois de nombreuses collectivités territoriales plusieurs milliers seraient concernés ont ainsi fait le choix de réduire, voire de supprimer l'éclairage public la nuit. On peut se féliciter de la conciliation de la sobriété énergétique des économies budgétaires et de la biodiversité. À ce titre je me permettrai observation qui ressort fortement des cartes de la pollution lumineuse. En France, il s'agit d'un phénomène avant tout urbain. Ce problème d'une France urbanisée est assez éloignée de celle que nous trouvons dans la plupart des départements les plus ruraux et les zones très peu denses. Une approche territoriale différencier de ce problème permettrait de mieux saisir des réalités distinctes éventuellement d'adapter les solutions locales. Si la France a développé une réglementation pour limiter les nuisances lumineuses. Il est aussi possible de voir dans cette nouvelle pratique un nouvel enjeu juridique pour le droit des collectivités territoriales. en effet. Le dans le. En effet le cadre juridique des décisions des élus locaux notamment des maires. Elle pose aussi le problème de la mise en cause de leurs responsabilités en cas d'accident ou de violence. Les nouvelles pratiques de l'éclairage public, nécessite ainsi je le pense, la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire. Au-delà de la jurisprudence existante. Le droit doit évoluer avec la pratique profondément transformé ces 2 dernières années afin de donner un cadre juridique clair aux élus locaux pour qu'ils puissent exercer leurs compétences aussi Madame la Ministre. Le gouvernement compte-t-il légiférer sur le sujet de la suppression ou de l'extinction de l'éclairage public. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci monsieur le le président, mesdames, et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur Englaro. En effet, le maire est chargé de la sûreté de la commodité du passage dans les rues. Qu'elle place et voie publique, ce qui comprend le nettoiement et l'éclairage cependant aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales, une obligation d'éclairage de l'ensemble des voix de de communication si le service public de l'éclairage extérieur revêtent un caractère obligatoire, il n'implique pas pour autant un droit d'éclairage pour l'usager ou le riverain d'une d'une voie publique, en revanche, le maire doit chaque fois qu'il qu'il a conscience, ou aurait dû avoir conscience d'un danger en vertu de son pouvoir de police signalé aux usagers les risques qu'ils rencontrent de nuit. L'éclairage public est loin d'être la, la seule solution pour sécuriser un endroit dangereux. Des mesures de signalisation visible de nuit tels que des panneaux réfléchissants ou clignotant avertissant des dangers ou encore les installations d'éclairage programmables ou pilotage à distance peuvent parfaitement suppléé à l'éclairage continue encore de nuit dans les fêtes, on note qu'il y a davantage d'accidents ou d'agressions en plein jour ou dans des zones illuminé à titre exemple il a, il y a plus de 2 cambriolages en plein jour. Autre exemple concernant la sécurité routière. Par exemple l'autoroute la la 15. N'est plus éclairée depuis 2010 et pour autant, aucune augmentation d'accidents n'est observée. Malgré le fait qu'il y ait plus de personnes à prendre à prendre cette cette voix, donc vous voyez bien que, que, en tous les cas ça ne se vérifie pas ce que je peux vous confirmer en tout cas, évidemment, c'est que la vie des mères et est extrêmement important sur sur ce sujet et qu'on sera évidemment vigilants à ce que soient pas quelque chose qui puisse. Nuire ou en tout cas être être difficile pour pour les élus. Merci. La parole est à monsieur Franck Menonville pour le groupe les indépendants pour 2 minutes. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Les astronomes ne sont pas les seuls à subir la gêne de la lumière trop forte ou mal dirigé ou mal orienté les méfaits de la pollution lumineuse ne sont pas non plus à démontrer tant pour la faune et la flore que pour nos concitoyens également. En matière de d'éclairage public cependant les intérêts doivent être concilié bien qu'il s'agisse d'une source majeure de pollution lumineuse, l'éclairage constitue également l'une des composantes de la sécurité et du confort de nos concitoyens des rues bien éclairés, sont souvent des rues plus sûres. À ses intérêts s'ajoute la nécessité de réduire notre consommation d'énergie en particulier nos collectivités dans un contexte de dérèglement climatique et de hausse des prix. Désormais nous voyons. Nous voyons des mesures de bon sens, notamment les commerçants éteindre leurs vitrines. À l'heure auquel personne ne circule pour faire. Ses emplettes ses courses et des boutiques de toute façon fermer. Outre la réglementation, la technologie doit aussi permettre de parvenir au au bon équilibre une expérimentation d'un autre d'un éclairage intelligent et autonome a ainsi eu lieu à Bordeaux. De même dans la ville du président Larché Rambouillet on teste un éclairage public bio luminescents. Dans ces 2 cas, il s'agit de solution développées par des sociétés françaises très innovantes. Sur la gestion de son éclairage public notamment. Il nous semble primordial que la France reste souveraine. Madame la Ministre des mesures sont-elles prises par le gouvernement afin de soutenir ses activités afin que notre pays ne développent pas de dépendance à des technologies étrangères en matière d'éclairage public de lutte contre la pollution lumineuse, quel levier, mobilisez-vous. Ah si cher collègue, madame la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur Menonville les technologies d'avenir concernant l'éclairage public sont les LED. C'est sur cette. Technologie que l'industrie française doit consolider sa place prédominante en Europe et aussi dans le monde, effet un fort intérêt pour les entreprises françaises à se positionner sur le développement des technologies intelligentes comme le pilotage de l'éclairage public en particulier de la reconnaissance d'objets au passage que soit des humains un animal ou encore un véhicule. Le but est de passer du radar qui ne fait que détecter un passage à proximité de l'éclairage public à l'acquisition d'images pour non seulement savoir quels objets passe mais également sa vitesse pour synchroniser l'allumage et l'extinction. Si le passage au LED permet de diviser par 3 la consommation énergétique. Ces nouvelles technologies permettrait de diviser la facture par six. Notre industrie a également développé une compétence reconnue à l'international dans la conception quasiment clés en main d'un parc luminaires. Il s'agit de répondre à la recherche d'une signature visuelle typique de nos collectivités mais également à une forte demande de rétro vite, c'est-à-dire le passage de la lampe classique à la LED sans modifier le Design du luminaire. Ce qui est intéressant pour nos entreprises françaises c'est la tête de la LED qui représente le composant le plus stratégique en revanche qui ne relève pas de de l'innovation, c'est-à-dire les plaques des LED qui ont une faible valeur ajoutée et le marché en plus Les industriels français ont aujourd'hui un vrai savoir-faire et une capacité à innover. Elles sont par exemple leader mondial en éclairage solaire. Donc c'est plutôt vers ça que je, j'amènerai les, les entreprises et les industriels français à à à mener leur projet. Je vous remercie. très négligée. Si on compare avec la lutte contre l'artificialisation celle-ci bien a raison est engagée, elle touche 3% des sols, la pollution lumineuse un pack tel 23% de la surface terrestre et ça vient des 10 85 % en France. Alors est-ce que c'est une pollution négligeable. si grave que ça, de ne pas pouvoir observer la Voie lactée. Il y a une chanson enfantine qui le dit fort justement la nuit c'est pas comme le jour c'est pas vrai, tout est différent. D'abord je ne vois pas ben ensuite on réapprend l'obscurité ensuite on tâtonne sous la voûte étoilée. C'est une des meilleures façons de se reconnecter à notre environnement de profiter du d'une appréhension sensorielle très riche du monde et de s'extraire. Comme le dit si bien la note de notre collègue Annick Jacquemet de s'extraire d'une vision anthropocentriste. S'ils disparaissent nous disparaissons. C'est le grand titre de Libé ce matin sur les insectes. Hé bien de la pollution lumineuse. Elle est responsable de la mort de milliers de milliards d'insectes. Alors depuis le Grenelle, on a entamé effectivement la lutte progressivement les textes se complètent mais où est l'efficacité en termes de résultats l'éclairage public, relève de l'action volontaire des collectivités. Est-ce suffisant, surtout qu'aujourd'hui l'avait demandé l'aide réduit le gâchis énergétique certes mais aggrave si on ne les pas bien la toxicité sur la biodiversité, la santé, il y a aussi encore des mangues, ça a été dit l'arrêté sur les seuils de l'imminence des publicités n'a toujours pas été publié. Un décret sur l'extinction des publicités et va entrer en vigueur. Avec le reste de de nos mesures normatives permettra-t-il de faire éteindre les dispositifs qui devrait légalement lettre on en est loin. Le contrôle est très rare les sanctions encore davantage. Comment l'État compte-t-il assurer l'application de la loi et enfin sur la biodiversité. Le cadre législatif et réglementaire terrestre très reste très léger. Êtes-vous résolue, madame la ministre a consacré à affermir la trame noire dans le code de l'environnement. Merci madame la ministre. ce n'est pas une pollution année 2 anecdotique et je vous remercie d'avoir rappelé un certain nombre de faits. Un constat qui est évidemment alarmant. Pour la biodiversité et particulièrement pour les insectes en France et en effet la première page pardon de Libé montre bien le le la la difficulté dans laquelle on est. Vous avez aussi raison sur le fait qu'il y ait des des décrets qui qui soit en retard et pour ça il faut que nous rappelions un petit peu la patrouille et que nous nous soyons à la hauteur. Moi ce que je peux vous dire aussi c'est que le fait de partager ce constat ce soir et d'avoir madame la rapporteure amener ce sujet en débat. Aujourd'hui aussi important parce que ça nous permet justement de rappeler tout ce qu'il nous reste à faire et de prendre aussi des engagements auprès de vous, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Directement dans mon propos introductif lorsque j'ai pris un certain nombre d'engagements. Le rapport de l'eau ne cesse avait mis d'ailleurs en avant le besoin de limiter l'utilisation aussi des, des groupes de risques. De étroit, c'est-à-dire les, les lettres qui ont une forte honneur en couleur bleue vous l'avez d'ailleurs cité madame la rapporteure. Et si dans le spectre de couleurs, c'est vraiment problématique. Et il faut que nous agissions là-dessus l'obtention de de certificats d'économie d'énergie sur les luminaires d'éclairage à modules LED imposent. Déjà des, des groupes de risque, 0 et 1 pour bénéficier du du CE et les industriels ont priorisé pour le luminaire destinée à l'éclairage public ces 2 groupes 0 et La révision de de l'arrêté du 27 décembre 2018 pourra être l'opportunité d'entériner la limitation au groupe de risque 0 et un pour les l'éclairage public et sur le paradoxe que vous mentionnez entre le gain énergétique et la protection de la biodiversité, à mon sens il n'y en a pas, au contraire, nous pouvons satisfaire les deux et en même temps, je vous rejoins sur la nécessité de créer des trams noir. En parallèle de ce qui sera prévu dans la prochaine SNB, je l'ai d'ailleurs aussi rappelé et des expérimentations sont en cours. Moi j'ai pu noter des propositions intéressantes dans le cadre de d'une discussion en commission développement durable de l'Assemblée nationale, c'était assez récent pour que je vous en parle. C'était le 29 mars dernier. notamment proposait que l'État puisse réglementer et restreindre les éclairages publics et privés en coeur de nuit pas restriction de la puissance lumineuse ou l'extinction il proposait également que l'État puisse mettre en place des aires de protection de la faune nocturne et du ciel étoilé par la création de tram noir dans les espaces protégés. Ce qui permettra donc un certain nombre de Français de retrouver le plaisir de regarder un ciel étoilé, il me semble intéressant que nous travaillons rapidement autour de ces idées sur lesquelles nous pourrions aller rapidement. Ça relève pas forcément d'un de discussion législative mais que ça peut être. Avancé dans le cadre réglementaire, donc je pense que nous pouvons avancer assez sereinement et rapidement sur ce sujet. Merci madame la ministre. La parole est à madame Nadège avait pour le groupe RDPI pour 2 minutes. que nous puissions débattre de la pollution lumineuse. À la suite de vos travaux, madame la sénatrice Jacquemet, une note a été. Rappelons que plus de 3 humain sur 10 ne peuvent voir la voie lactée la nuit. Ça monte à 6 sur 10 en Europe et à 8 sur 10 aux États-Unis, en France, le nombre de points lumineux a augmenté de plus de 50% en 30 ans un phénomène de très grande ampleur directement imputables à l'activité humaine dont on parle moins que d'autres. Cet état de fait a comme conséquence des nuisance sur la faune et la flore sur leur cycle perturbé par cette illumination perpétuelle du ciel, les oiseaux migrateurs, les insectes et les chauves-souris sont les espèces les plus touchés, alors qu'elle joue un rôle central en matière de biodiversité. En 2018, un arrêté relatif à la prévention à la réduction à la limitation des nuisances lumineuses est venu encadrer les installations d'éclairage public et privé pour réduire leurs incidences sur la biodiversité, plus récemment la COP15 biodiversité de Montréal a abouti à un accord. Les cibles de et sept qui figure viennent traiter de la restauration des écosystèmes dégradés et la réduction des pollutions à la source notamment lumineuses les trams noirs ont été intégrées à la stratégie nationale biodiversité 2030 ces corridors écologiques d'obscurité constitue un véritable une véritable respiration pour des écosystèmes fortement perturbé Roubaix c'est. Ces dernières décennies. Madame la Ministre, quelle évaluation faites-vous de l'application de l'arrêté de 2018 et de ses effets dans la stratégie nationale biodiversité quelles actions sont déjà mises en Oeuvres dans le cadre du volet incitation au développement des trams noirs et les intentions en matière de lutte contre la pollution lumineuse. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci monsieur le le président, mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice avait l'arrêté du 27 décembre 2018, fixe des obligations aussi bien. En temporalité qu'en termes d'exigences techniques. Le contrôle est du ressort du maire sauf pour les installations communales pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État aujourd'hui, soyons très clairs. Les contrôles de cette réglementation sont insuffisants. J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis parce que je pense qu'il faut que nous agissions. Dans mon discours d'introduction, je je je vous ai dit souhaiter travailler sur la mise en place d'une amende forfaitaire. Type carnet de souche pour simplifier la prise de sanctions sans avoir besoin d'une décision nécessitant l'appréciation du juge. Où est la poursuite au préalable du parquet. Ensuite, nous souhaitons également cibler les contrôles sur la pollution lumineuse, réalisé par l'OFEV dans les zones les plus sensibles pour la biodiversité. Ce sera dans la stratégie nationale biodiversité et enfin le Centre scientifique et technique du bâtiment travaille sur une méthodologie simple et pratique pour permettre le contrôle de la partie technique de la réglementation. Il s'agit par exemple de la vérification de la température. De couleur, de la part de de lumière émise au du de l'horizontale de l'intensité lumineuse. Voilà le le temps me manque pour détailler ce qui sera prévu dans, dans le second volet de la SNB je prendrai plus de temps pour vous répondre précisément sur ce point je suis certaine qu'on aura l'occasion de, d'en reparler juste après. Si madame la ministre. La parole est à monsieur Joël Bigot pour le groupe socialiste, écologiste républicain pour 2 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, aujourd'hui un tiers de l'humanité ne peut plus distinguer la voie lactée la faune, la flore, la font je sont affectés par la pollution lumineuse. Les animaux diurnes et nocturnes voient leur cycle de prédation détériorée au détriment de la chaîne alimentaire. Le sur-. Éclairage est également la 2ème cause de mortalité des insectes. Après les pesticides le rythme circadien humain est également déstabilisé, entraînant de nombreux problèmes de santé pour l'homme. Le constat est alarmant, les progrès en matière de performance de d'éclairage sont assorties d'un effet rebond qui conduit à un élargissement des zones éclairées à hauteur de 2% annuels dans le monde aussi. La technologie LED et pourfendu par les associations qui dénoncent l'augmentation de la lumière bleue plus dangereuse pour la biodiversité. Quand le rapport de l'Opecst relativise le bilan carbone de nombreuses solutions existent d'abord à droit constant, il faut faire respecter l'arrêté du 27 décembre 2018 qui encadrent l'éclairage privés mais dont les associations relève la non application en fait. En Maine-et-Loire, France Nature Environnement et la Ligue de protection des oiseaux sont particulièrement active elle recense les lieux d'éclairage potentiellement illégaux et sensibiliser les acteurs privés comme les collectivités, malgré un coup d'intervention du syndicat de l'énergie des communes d'Anjou sont volontaires pour dans des politiques d'extinction à Saumur des Russes ont équipé depuis 8 ans de réverbères avec des cellules qui détectent les voitures et piétons permettant d'économiser près de 90.000 euros pour une commune de 27.000 habitants dans ce même département, le Centre permanent d'initiatives environnementales Loire Anjou accompagne les communes dans l'élaboration de tram noir en identifiant les zones à enjeu pour la biodiversité. Une bonne pratique identifiés par le rapport de l'Opecst Madame la Ministre quels engagements prenez-vous pour accompagner ces initiatives locales et concrètes et assurer les politiques publiques de l'État et dans l'initiative réglementaire, la promotion des solutions partout en France pour retrouver la nuit je vous remercie. moi je partage votre constat sur l'impact très important de la position lumineuse sur la biodiversité. Vous savez à quel point ce sujet me me tient à coeur, surtout dans un contexte où nous venons d'aboutir à un accord mondial lors de la COP15 qui sera repris, notamment dans la stratégie nationale biodiversité qui sera annoncé prochainement votre question enfin votre question en tout cas votre. Un certain nombre de constats que vous avez fait et puis les les questions que vous avez posées permettent de de de détailler ce que nous prévoyons justement dans la SNB pour lutter contre la pollution lumineuse et préserver notre biodiversité, je souhaite vous partagez 4 actions. La première c'est d'améliorer la connaissance des impacts de cette pollution sur la biodiversité, grâce à de nouveaux indicateurs à l'enrichissement des bases de données via notre observatoire, c'est également d'éviter les impacts des équipements lumineux en améliorant le Conseil des distributeurs auprès de leurs clients. Et également, de développer les trams noirs dans les territoires. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas être enfin peut être plus plus exhaustif sur ce sujet et enfin comme j'ai dit précédemment aussi c'est de mieux cibler une partie des contrôles sur les espaces les plus sensibles pour la biodiversité comme vous moi je souligne, ce qui a pu faire la la la ville de Saumur qui a fait ça il y a maintenant plusieurs années alors qu'on parlait assez peu de ce sujet jusque-là et dire évidemment que le fond Vert accompagne les collectivités dans cette, dans cette prise d'initiative. Ça a très bien marché, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de projets qui portent sur les éclairages publics et c'est tant mieux. Je pense qu'il faut. Évidemment continuer dans ce sens et nous avons bon espoir avec Christophe Béchu de pérenniser le Fonds Vert pour que ça puisse continuer à accompagner les collectivités dans ce sens. Merci madame la ministre. La parole est au président Jean-François Longeot pour le groupe Union. Merci monsieur le président, madame mise, mes chers collègues. La pollution. Est multi-face et multi-facettes les déchets le carbone, les transports pollue. Mais la lumière aussi pour la pollution lumineuse est l'une des grandes oubliées des politiques environnementales. Si vous me passez l'expression, nous ouvrons à peine les yeux dessus. C'est pourquoi la note que vient de publier l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le sujet, si précieuse. Je tiens en particulier a su élever le travail de ma collègue du Doubs Annick Jacquemet qui en est l'auteur. C'est la première fois que le Parlement s'intéresse au phénomène. La première fois qu'il en établit les caractéristiques, les effets et avance des solutions pour y remédier. Parmi les outils dont nous disposons aujourd'hui à l'échelle locale pour passer d'un éclairage systématique à une adaptation fine de celui-ci selon contexte pour reprendre les termes de la note de l'Opecst figure le Fonds Vert. Il a officiellement été ouvert en janvier dernier sous forme d'un guichet unique pour les collectivités. Doté de 2 milliards d'euros, il a vocation à subventionner à hauteur de 40%. Les projets de transition écologique des collectivités. Parmi ces projets de transition figure la rénovation des éclairages publics. Une remise pris des premiers Aurélia lauréat a eu lieu la semaine dernière, avec des résultats encourageants puisqu'au total les projets déposés depuis janvier ont atteint l'enveloppe de de des 2 milliards d'euros de subventions. D'après nos informations, vous pourrez. Nous le confirmer. Madame la Ministre les ai visiter des projets en cours d'étude. D'après nos informations toujours beaucoup d'entre eux concerne justement l'éclairage public. Combien. Et en quoi consistent ces projets et vont-ils servir à lutter contre la pollution lumineuse. Objet du présent débat je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, monsieur le le président l'Anjou. Annoncée par là. Première ministre le 27 août dernier le Fonds Vert doit permettre le déploiement d'action territorial de, de transition écologique. Il a été ouvert officiellement. En janvier dernier sous le pilotage des préfets et sous forme de guichet unique pour que la démarche des collectivités, soit la plus simple possible et c'est un vrai succès puisqu'à l'heure où je vous parle, les dossiers déposés ont été très nombreux, environ 7000 et l'enveloppe dédiée de 2 milliards d'euros a été atteinte. Les dossiers sont actuellement en cours d'étude. Ça veut pas dire que les 2 milliards d'euros ont été dépensés. Je, j'insiste parce que ça veut dire que vous pouvez continuer à inciter les territoires a déposé évidemment des projets. Concernant la rénovation énergétique et et l'éclairage public. Ils ont eu le succès le plus rapide hein. Dans le cadre de ce fonds Vert, c'est une bonne nouvelle pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui car accélérer la la rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public. C'est un moyen de lutter contre la pollution lumineuse. Le Fonds Vert s'applique à l'éclairage public extérieur sécurisant les cheminements des personnes, il permet de financer des études comme un diagnostic territorial une stratégie d'extinction encore de nuits ou encore une création de tram noir ces subventions permettent à la fois de financier de l'ingénierie et surtout des investissements de modernisation du parc de luminaires. L'objectif est de diminuer le nombre de points lumineux et de baisser l'importance de la puissance, c'est un vrai levier pour accompagner les collectivités dans la dépollution lumineuses aujourd'hui 2000 projets concernent le renouvellement des des parcs d'éclairage public, soit 28% des projets déposés dans le cadre du Fonds Vert. Et par ailleurs nous nous étions fixé un objectif de rénovation de 10% du parc du parc d'éclairage je peux d'ores et déjà vous dire qu'avec les dossiers déposés nous atteindrons cet objectif je profite d'ailleurs de votre question, pour vous rappeler OK rappeler aussi que 150 millions d'euros du fonds verts sont dédié à la biodiversité. Cette enveloppe par contre n'est pas atteinte et donc je vous encourage vraiment à communiquer au maximum sur cette possibilité de subventions auprès des collectivités que vous représentez chacun je vous remercie. Merci, madame la Ministre, la parole à Monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues. Effondrement de la biodiversité, destruction des populations d'oiseaux et d'insectes allô lumineux ou du sud, des villes altérations du sommeil, augmentation des risques cardiovasculaires de cancers. On ne compte plus aujourd'hui les effets nocifs de la pollution lumineuse sur la santé du vivant des humains et aussi de notre environnement. Il fait d'ailleurs très bien documenté par de nombreuses études scientifiques. La croissance démographique doublée d'une forte urbanisation a conduit à l'explosion des émissions lumineuses notamment avec l'éclairage public. En plus de participer au dérèglement climatique en perturbant les écosystèmes cet éclairage artificiel nocturne contribue au gaspillage énergétique. Selon l'Ademe l'éclairage public correspond à 41% de la consommation d'électricité des communes. Et émet annuellement 670.000 tonnes de CO2. Afin de lutter contre ses nuisances lumineuses. La France s'est dotée d'une réglementation ambitieuse, selon les termes de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans une note datant de janvier 2023. Cette réglementation fait notamment du maire l'autorité compétente pour s'assurer du respect des dispositions de sobriété, de l'éclairage public nocturne. Je voudrais redire ici combien l'action à l'échelle communale est importante pour agir efficacement contre la pollution lumineuse dans mon département de la Mayenne, les élus sont conscients de ces enjeux et prennent des engagements forts, par exemple, la commune de La Bazouge des Halles a reçu le Label Village étoilés créé par une association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement et luttent activement pour la qualité de la nuit. De nombreuses communes de mon territoire, à l'instar de mon Jean se lance dans la révision de leur éclairage public en partenariat avec le syndicat territoires d'énergie Mayenne et d'ici 2026 tous les luminaires qui éclaire totalement ou partiellement vers le ciel doivent être remplacés ma et câbles compris pour les plus anciens pour la Mayenne, le coût de l'opération total s'élève à plusieurs millions d'euros. Donc à travers le Fonds Vert, entre autres, l'État peut accompagner utilement ce partenariat entre communes et le syndicat énergie. Il est nécessaire d'améliorer les critères d'éligibilité pour en collège fluide de cette coordination, je termine monsieur le président. et une réglementation qui est encore incomplète, comment le gouvernement compte accompagner encore plus nos territoires ruraux pour lutter contre la pollution lumineuse. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le le sénateur, je Chevrollier. J'ai, j'ai pu le le le dire déjà précédemment, mais nous souhaitons mieux accompagner les les collectivités dans leur lutte contre les pollutions lumineuses et le Fonds Vert pour le volet financement et la forfaitisation de l'amende pour le volet facilitation du contrôle accompagner les collectivités, c'est aussi les soutenir dans leur ingénierie. La formation et la formation des élus seront un chantier que le ministère devra ouvrir avec la révision de l'arrêté du 27 décembre 2018 en complément on les professionnels de de l'éclairage, les services de l'État et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies pourront être force de propositions pour aider justement les collectivités à faire le bon choix techniques concernant la mise en avant des collectivités vertueux tient à rappeler le soutien que le ministère accorde à l'association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturnes, en particulier pour son concours Villes et villages étoilés, vous l'avez d'ailleurs cité qui s'est étendu récemment au territoire. De même, le ministère à travers les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux soutient les territoires et les aide à porter des projets de réserve internationale de ciel étoilé, je vous remercie. Merci, madame la Ministre, la parole à Madame Martine Filleul pour le groupe socialiste, écologiste républicain pour 2 minutes. monsieur le Président Madame la Ministre, chers collègues, les élus locaux se mobilisent déjà depuis plusieurs années sur le sujet de la pollution lumineuse, leur approche sont multiples dans mon département doué, a mis en place une trame sombre avec une baisse de 90% de la lumière la nuit et des détecteurs de présence pour les humains. Lille afin de protéger ces corridors écologiques remplacent les anciennes LED à lumière blanche ou bleue qui représente une catastrophe pour la biodiversité par de nouvelles LED ambrées dont la longueur d'onde, ne gêne plus les espèces animales systématiquement les résultats sont éloquents. Aussi ces mêmes aspects néfastes sur les espèces animales sont également largement documenté sur l'être humain. Comme le souligne le rapport de l'Opecst se sont altérations du sommeil, trouble de la mémoire de l'humeur de la tension risque cardiovasculaires, cancers, diabète ou obésité. Oeuvrer dans ce sens pour une adaptation de l'éclairage privés et publics vers des LED de nouvelle génération, c'est agir pour la biodiversité et directement pour la santé de nos concitoyens. Madame la Ministre quelles orientations le gouvernement prévoit-t-il de prendre en la matière pour la santé de nos concitoyens. Entendez-vous compléter la législation pour lutter contre les risques de photos toxicité de certaines sources lumineuses, l'État a-t-il répertorier les bonnes pratiques mises en place par les élus locaux sur le territoire. Je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice filleul déjà je vous remercie de pour le partage de bonnes pratiques, vous avez cité certaines villes certaines communes qui qui participent justement à la à la dépollution lumineuses et je pense qu'il est toujours très intéressant de les citer parce que évidemment c'est intéressant de s'en inspirer Et moi j'ai déjà pu le. Le dire. Il y a certaines collectivités qui mettre en place un certain nombre de choses et je pense que c'est très intéressant qui l'équilibre des éclairages fasse l'objet d'une concertation avec les habitants de la ville de manière à répondre au mieux à leur usage de l'espace public. Vous avez raison, nous devons aller plus loin. Concernant les mesures que nous demandons. Aux différents acteurs. À ce titre, moi je me réjouis de la signature. Je l'ai dit le 27 mars dernier de la charte d'engagement des acteurs du du transport avec le ministère de la transition énergétique et de la transition écologique pour tendre vers plus de sobriété énergétique. Via des mesures d'extinction des panneaux lumineux. J'ai pu dire également que je souhaite que nous allions plus loin, en renforçant l'extinction des bâtiments non résidentiels actuellement leur d'extinction, s'étend de une heure à 7h du matin je souhaite une extinction plus grande et je prends l'exemple d'une du du d'une extinction à partir d'une heure après la fin de l'activité et une heure avant la reprise de l'activité. Je souhaite aussi que nous réfléchissions à la diminution des diminutions des nuisances lumineuses issus des serres et des verrières tels que les serres agricoles les éclairages excessifs et non directive de certaines ont des conséquences importantes sur la faune, les insectes, les oiseaux ou encore les chauves-souris ou aussi sur le paysage nocturne, on parle de ciel rouge et jaune. Je pense que nous pouvons aussi travailler sur la diminution des puissances lumineuse des stades avant et et après les événements sportifs, toutes ces mesures ne nécessite pas ne nécessite pas encore un véhicule législatif on peut agir aussi assez rapidement par voie réglementaire, je n'oublie pas les, les mots employés aussi par Madame la rapporteure notamment sur le sujet de la lumière bleue. Il y a eu notamment un rapport qui a été rendue sur justement la nuisance des des lumières bleues pour les enfants et je pense que il y a un certain nombre de choses que nous pouvons nous vont mener ensemble, réfléchissons. Avec évidemment ce que vous avez proposé dans le cadre de votre rapport également ce que vous pourriez être en mesure de proposer Mada fièvre. La parole est à madame Marie-Pierre Richer. Pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, je pose ma question au nom de ma collègue Martin décidera qu'à laquelle bien sûr je m'associe, en effet, on l'ignore mais pour près de 60% des Européens et 80% des Américains, il est impossible de pouvoir observer la Voie lactée. C'est environ un tiers de l'humanité qui est victime de ce que l'on appelle la pollution lumineuse qui touche également la biodiversité sur près de 20% des Terres émergées. De 1990 à 2010 les zones illuminés ont progressé de 6% par an le rythme reste aujourd'hui soutenu à peine tempérée par les récentes prises de conscience. Inéluctablement nos espaces de vie sont gagnés par la pollution lumineuse générant stress, anxiété et perturbations du sommeil ce phénomène exerce aussi une forte pression sur la biodiversité, avec des conséquences multiples dont certaines sont encore mal évaluée. Une telle perturbation du vivant ne sera pas à terme sans conséquence. Je pense notamment aux insectes essentiels au bon maintien des raisons tropiques. Dans de nombreuses communes, notamment celles de nos territoires. Des mesures ont été prises pour être un d'éclairage public aux heures creuses de la nuit à la maîtrise de la consommation énergétique préconisé dans le PC a été s'ajoute donc la protection de la digue là de la biodiversité, madame la Ministre, il nous faudra malgré tout aller plus loin pour atteindre un équilibre entre préservation de la biodiversité et progression des zones illuminé. Quelle feuille de route le gouvernement qu'on ne suivent pour y faire face. Sous quel délai, merci. l'équilibre entre préservation de la biodiversité et la progression des zones illuminé se trouve dans la multiplicité des solutions et le développement des technologies, la lutte contre les nuisances lumineuses peut en effet prendre diverses formes. Il y a évidemment l'extinction totale en coeur de nuit comme dans l'intégralité des communes du parc naturel régional du Gâtinais français. Mais cela peut aussi passer par le pilotage intelligent de l'éclairage, comme cela a été testé à Paris Bordeaux ou encore Toulouse. Cela doit être étudiée au cas par cas selon la volonté locale que ce soit pour la création de 3 femmes noires ou de réduction du halo lumineux des grandes métropoles, les solutions techniques existent et les leds ont cet Avantage de pouvoir avoir leur puissance moduler et gérer à distance aujourd'hui les collectivités rurales comme urbaines peuvent trouver une solution adaptée. Je vous remercie. Merci. Oui une réplique. Merci madame la ministre, on parlait autrefois avec admiration de New York comme la ville qui ne dort jamais. Aujourd'hui c'est l'inverse vers lequel nous devons tendre les maires en sont les acteurs essentiels. J'ai bien entendu vos mesures. J'espère sincèrement qu'elles produiront leurs effets, la protection du vivant et notre qualité de vie sont à ce prix pour les générations d'aujourd'hui à vous. Merci, cher collègue, Monsieur le questeur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste, écologiste républicain pour 2 minutes. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre j'ai. Vu que vous parliez de la charte et alors j'ai été très impressionné par un article qui a été fait par monsieur Stéphane. Foucart dans le journal Le Monde. Je pense qu'il ne vous a pas échappé. Et alors il dit qu'il est dit dans cette charte qu'il faut équiper progressivement les dispositifs de publicités lumineuses afin que ceux-ci puissent être éteints. Très bien. Qu'il faut mettre en oeuvre lors de la fermeture des gares, stations, aéroports, l'extinction ou la mise en veille des publicités lumineuses équipée du dispositif le permettant. Et si le dispositif ne le permet pas, naturellement, il se passe rien. Et puis alors il y a ce chef-d'oeuvre vraiment je félicite l'auteur, vous le connaissez peut-être Madame la Ministre on nous parle d'établir une stratégie sobriété fondée sur des trajectoires de réduction de consommation électrique et d'émissions carbone du parc des publicités lumineuses en tenant compte des caractéristiques usage et besoins des univers de transport selon leur périmètre à la date. Vous rendez compte, en tenant compte des conditions du contexte et du périmètre. Tout ça n'est pas très. Claire. Le moins qu'on puisse dire c'est que c'est vague et flou. Alors ma première question c'est consiste à vous demander si vous allez muscler un peu tout cela. J'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure mais il ne faut pas qu'on en reste au niveau des intentions et comme il reste encore quelques secondes. Je voulais vous demander ce que vous comptiez faire particulièrement pour les publicités dans les entrées de ville. Les entrées de ville sont un gros problèmes urbanistiques. On a fait des catastrophes dans toutes nos agglomérations avec des entrées de ville qui ne sont pas très urbaine. Et voilà que l'on a des publicités énormes. On ne voit qu'elle, on ne voit que la publicité à toutes les heures de la soirée et même de la nuit. Donc, que comptez-vous faire pour mettre fin à cette pollution pollution totalement inutile et qui est préjudiciable. Monsieur le président. Merci. Merci monsieur le le président, mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur sueur. Vous dire évidemment que je n'ai pas échapper à la lecture. De l'article du Monde. Sur justement la charte qui a été signé. Et qui a été initiée notamment par Clément Beaune et Agnès Pannier-Runacher. Moi j'ai été très clair dans ma prise de parole, j'ai rappelé que les opérateurs s'étaient engagés s'était engagé à éteindre 100% de leurs panneaux lumineux dès la fermeture des gares, des aéroports et des métros. D'ici au 1er janvier 2024. Il s'engage également établir une stratégie de sobriété, de la gestion de leur parc de panneaux lumineux la RATP s'est engagée à réduire sa consommation électrique d'ici 2026 de 35% la SNCF de 45% d'ici 2031 et ADP de 50% d'ici 2030. Moi je crois que. Au-delà des incitations ou même des obligations légales. Je pense que il faut aussi faire confiance à des heures opérateur aussi important en France. Des opérateurs qui ont pris des responsabilités à un moment on a aussi une parole politique je viens la confirmer ici ce soir dans le cadre de ce débat organisé au Sénat. Je crois que c'est important aussi de de noter que la le politique peut avoir du poids, on verra comment les engagements sont suivis. Moi je suis très curieuse de voir comment la RATP va réduire justement sa consommation électrique d'ici 2026. Mais on ne va suivre ça de près. Des engagements ont été pris et je crois que il faut faire confiance aussi à des opérateurs, encore une fois qui ont pignon sur rue, on parle d'opérateurs de transport qui sont des opérateurs importants avec qui on a des discussions qui sont très régulière, vous m'avez posé une question plus précise concernant les, les, on va dire le la publicité lumineuse particulièrement sur les entrées des communes. Sachez qu'il y a des évolutions réglementaires qui sont en cours d'élaboration. Déjà un projet d'arrêté qui permettra de fixer des normes techniques applicables aux publicités lumineuses. Également un projet de décret qui permettra de limiter le format des panneaux d'affichage extérieur et son objet est plus large que la seule publicité lumineuse. Mais il s'appliquera à la publicité lumineuse et aussi non lumineuses. Ça c'était un décret qui est en attente. Je m'en charge. Et je vais m'en occuper pour qu'il sorte rapidement.

monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. C'est un cauchemar, je ne vois plus la Voie lactée et comme compte je ne peux plus méditer sous le ciel étoilé. Voilà un exemple de cette pollution lumineuse qui nous prive de certains trésors de la vue qui sont, en fait, ceux de l'esprit. La lumière artificielle nocturne s'est beaucoup répandu. Elle ne cesse par ailleurs d'augmenter dans le monde. Dans un contexte de hausse des coûts de l'énergie aussi bien pour les collectivités que pour les individus. La lutte contre la pollution lumineuse est une nécessité. Sur le plan de la santé. Elle a fait que nos écosystèmes elle perturbe aussi les équilibres écologiques comme la perte d'orientation des oiseaux migrateurs. Les nouvelles technologies ont apporté des solutions. Il y a des ces éclairage intelligent mais aussi ceux qui depuis quelques années, ni le même plus le ciel mais la rue enfin sans impact sur l'environnement naturel. Beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire. Alors, ne tombons pas dans une, dans un autre extrême en passant de la pollution lumineuse à l'obscurité intégral la lumière c'est une maîtrise par l'homme, de son environnement. La lutte contre la pollution lumineuse doit être un vrai progrès collectif et non une énième démarche punitive un combat au service de tous et non une futile initiative qui oppose les uns aux autres. Madame la Ministre beaucoup de questions sont posées, on a vu le sujet est très large car ce combat demande de nombreuses actions et surtout un vrai pilotage des expérimentations ont eu lieu dans certaines zones protégées quelles leçons peut-on tirer de ces dispositifs doit-on les généraliser. Qu'en est-il de la cartographie de ces expérimentations. Et que comptez-vous faire pour accompagner les collectivités locales et lutter contre cette pollution lumineuse, les aider à choisir les techniques les plus efficaces nos communes doivent être aidés dans l'ingénierie et dans les investissements et réellement compenser enfin comment mieux protéger cet environnement nocturnes. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Dans le temps que j'ai pour vous répondre, je vais me focaliser sur votre question concernant les expérimentations les aires protégées sont d'excellents territoire pour expérimenter de nouvelles approches en matière d'éclairage ces espaces abritent souvent des enjeux de préservation de la biodiversité nocturne et bénéficie d'instance de concertation qui permettent d'avancer collectivement sur ces sujets, on peut citer par exemple l'action des parcs nationaux. Comme le parc national des Cévennes, cité par madame la sénatrice Pentel tout à l'heure, c'est pas et, par ailleurs, un exemple de mobilisation d'acteurs multiples. Des équipes du parc national, les élus, les habitants les partenaires institutionnels, également les syndicats d'éclairage, de la Lozère et du Gard, les parcs naturels régionaux sont aussi des territoires actif et précurseurs. Ils peuvent réduire l'éclairage public nocturne comme le PNR Gâtinais français a pu le faire, je l'ai déjà. Indiqué plusieurs actions tourné vers la maîtrise de l'énergie ont conduit notamment à l'extinction de de l'éclairage la nuit pour la majorité des communes du parc également ils peuvent rénover le matériel vétuste d'éclairage public avec le financement de projets innovants alliant sobriété énergétique, réduction de la pollution lumineuse et de l'impact sur la biodiversité. Cela a été mis en place par le PNR des causes du du Quercy et également le PNR Préalpes d'Azur. Je souhaite que nous généralisons. Cette démarche dans tous les parcs nationaux et régionaux, j'en ferai part aux responsables de de ces parcs. Je vous remercie. Merci madame le Ministre, la parole est à monsieur Marc Laménie pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci monsieur le président, madame la ministre. Madame la rapporteure et merci. pour. L'engagement de ce débat de qualité sur la pollution lumineuse au titre de. un des, beaucoup de questions ont été abordées. Beaucoup de sujets. Je voudrais pas faire de répétition mais c'est vrai que qui intéresse je dirais toutes et tous. Le volet collectivités territoriales a été aussi largement engagé. Je prends le département des. Ne sans le vouloir j'succède à ma collègue du même département. Il y a 449. Communes. Bon beaucoup de de villages de Bourg. Et. Également bon beaucoup ont.

De ce côté. Alors vous avez abordé je dirais le le financement des économies d'énergie, les fédérations départementales. Les syndicats d'électrification les collectivités locales. S'engage aussi pour investir pour économiser et je crois que c'est réellement important donc. Ma question c'est un petit peu l'articulation. Le Fonds Vert, vous en avez, vous en avez parlé mais il y a également aussi la la DETR la déciles. Il y a aussi d'autres financements au niveau de l'État. Je vous remercie beaucoup. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le le sénateur Laménie j'ai pu l'évoquer précédemment mais en effet il faut le rappeler le fond Vert. Il représente un accompagnement financier pertinent et efficace pour les collectivités territoriales. En revanche, nous devons désormais réfléchir à la montée en puissance justement de ce type de dispositif pour accompagner encore plus. Les collectivités dans leur lutte contre la pollution lumineuse et les économies d'énergie et vu la part des dossiers déposés visant à rénover le parc d'éclairage public. On voit l'envie. Le besoin des collectivités qui se confirme et vraiment on ne peut que se réjouir au sein de du ministère de la transition écologique. En charge également de la cohésion des des territoires. Pour cette raison, des réflexions sont actuellement en cours. Notamment pour pérenniser le fonds en 2024. Dans ce cadre, nous pourrions réfléchir à des critères spécifiques de préservation de la biodiversité pour octroyer des aides au renouvellement du parc d'éclairage public et d'autre part d'orienter certains projets qui ont été déposées dans le cas de du vers, vers d'autres enveloppes existantes et dont le plafond n'a pas encore été atteint. L'objectif est bien de pouvoir financer d'autres projets dans le cadre du Fonds Vert et donc probablement d'autres projets de rénovation d'éclairage public, je vous remercie.

Merci cher collègue. Enfin, la parole est à madame Laurence Muller-Bronn pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors ce débat nous donne l'occasion de revenir sur le sujet essentiel de l'éclairage public pour les collectivités locales et bien entendu sur l'importance des factures énergétiques le budget global la conversion des parcs lumineux vers des systèmes innovants de l'aide est non seulement indispensable mais urgente aujourd'hui 40% des installations d'éclairage ont plus de 25 ans et sont particulièrement polluante et énergivores. C'est un gain immédiat pour les finances communales puisqu'elles peuvent gagner jusqu'à 80% d'économies sur leur facture énergétique. Nous l'avons aussi entendu c'est un gain pour l'environnement pour la biodiversité et pour la santé humaine. Contrairement à d'autres investissements de moyen et long terme. Le gain énergétique et environnementale d'une conversion accélérée du parc sur le territoire serait immédiat. Pourtant, ces projets, vous l'avez dit Madame la Ministre représente 28% des crédits alloués par le Fonds Vert, on peut s'en réjouir, mais pour moi ça me semble trop peu selon les chiffres qui ont été communiqués par vous et par la Première ministre de la semaine dernière. Pourquoi madame la ministre, avoir choisi d'intégrer les subventions à l'éclairage public dans ce fonds Vert en concurrence avec d'autres projets alors qu'il y a urgence à éclairer mieux pour réduire les nuisances évoqué ce soir ce potentiel immense de rénovation, dont les bénéfices sont immédiats aurait dû être prioritaire, il serait déjà bien engagée. À l'heure où nous avons ce débat. Merci cher collègue. Madame la ministre. la phase d'instruction des dossiers déposés dans le cadre du fond Vert est en cours et un des critères exigés par l'État. Et l'impact écologique du projet, autrement dit les subventions seront octroyés pour des projets qui ont une réelle efficacité dans la transition écologique. C'est un point d'attention majeure qui fait toute la crédibilité bien sûr du Fonds Vert et qui nous permettra d'avoir la crédibilité de pouvoir en avoir aussi pour 2024. À titre d'exemple, environ 20% des dossiers déposés pour la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux déclare un gain énergétique inférieure à 30% qui est le minimum cité. Pour l'éligibilité avec même un objectif national de 40% de gains en dessous du seuil, cela ne peut être éligible au fonds Vert, même si les dossiers, on peut être leur intérêt par ailleurs pour l'éclairage public. L'objectif était de rénover, plus de 10% des parquets existants et de baisser les consommations électriques. Comme j'ai pu le dire précédemment cet objectif de 10% est atteint par les dossiers déposés. Je m'en réjouis. Par ailleurs, je peux d'ores et déjà vous dire que les projets de rénovation. Du parc d'éclairage public pourrait représenter 414 millions d'aide pour un milliard d'investissements, si tous les dossiers sont financés, cela représente tout de même près d'un quart de l'enveloppe globale permettra de rénover un million de points lumineux sur les 4 millions de points lumineux déclarés par les collectivités comme devant être rénovées. Donc, je crois pouvoir dire que c'est un succès et je pense qu'on peut s'en réjouir. Merci. Merci madame la ministre, une réplique Madame Muller-Bronn. Oui alors ce nouveau fonds ouvert pour les collectivités territoriales, est en réalité un recyclage des crédits du programme 362 on passe juste une gestion centralisée à une gestion pseudo décentralisé un plan national ambitieux avec un guichet unique pour l'accompagnement de l'ensemble des projets aurait sans doute été plus efficace, plus rapide et plus appréciée par les, les élus locaux, sur leur prochaine facture d'électricité. Merci. Merci cher collègue donc. Tous les intervenants ont pris la parole. Il reste maintenant pour conclure madame Annick Jacquemet au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour cinq minutes. minutes. Oui c'est mieux. Monsieur le Président Madame la Ministre Mesdames et messieurs les sénateurs. À l'issue de ce débat, je constate avec satisfaction qu'il se dégage un consensus au sein de notre assemblée pour lutter contre la pollution lumineuse. J'ai entendu vos propositions Madame la Ministre. Concernant la forfaitisation des sanctions sous forme d'amendes. La réduction des périodes d'éclairage intérieur des bâtiments, la généralisation des trams noirs dans les espaces protégés ou encore l'engagement volontaire des gares et des aéroports pour limiter les publicités lumineuses. Néanmoins je n'ai pas obtenu toutes les réponses aux questions que je vous avez posé hein si vous ne nous avait pas précisé quand tu l'arrêté fixant les seuils maximaux ne limitant. Des enseignes et des publicités et des publicités seraient enfin publié et surtout quelles seront ses grandes lignes. Par ailleurs, vous avez soutenu l'extinction de l'éclairage au corps de la nuit Monsieur Anglade comme moi même avons souligné la responsabilité qui pèse sur le maire en cas d'accident. Vous avez dit qu'il y a pas d'obligation générale à l'éclairage. Toutefois, il semblerait que la jurisprudence fait la distinction entre la situation où il n'y a jamais eu de lumière dans ce cas la responsabilité du maire n'est pas engagé. En revanche, lorsqu'il y avait. Éclairage et que le maire décide de l'éteindre. Il semblerait que sa responsabilité soit engagée. J'insiste donc sur le fait qu'il faudrait changer cette règle pour ne pas compromettre les initiatives des mères pour une plus grande sobriété lumineuse. Autre question sur les trams noir au cours de mes auditions m'en fait remarquer que ces dernières ne figure pas dans le code de l'environnement, ce qui les rendrait fragile juridiquement. Faut-il donc les cités dans ce code de l'environnement. Enfin, vous n'avez pas répondu sur les engagements pris dans le 4ème plan santé-environnement notamment en ce qui concerne les phares des voitures. Comme vous l'avez souligné 2 types de mesures doivent être prises, il faut d'abord compléter la réglementation et la faire respecter. À cet égard je souhaite faire une proposition de loi sur le sujet. Eh bien noté votre intérêt pour la pollution lumineuse et votre volonté de travailler avec le Sénat. Donc, c'est avec plaisir que nous continuerons à développer ce dossier, il faut également éduquer et sensibiliser nos citoyens et en particulier les plus jeunes au cours de mes auditions j'ai été marqué par les propos des responsables de l'Association française d'astronomie, qui constatait que le ciel est Toyer et le ciel étoilé avec l'émerveillement qu'il suscite, reste l'un des rares spectacles gratuits à la portée de nos concitoyens. Pourtant, une grande partie d'entre eux en sont privés. Ça a été relevé plusieurs fois ce soir avec un risque de déconnexion croissante des individus et des sociétés de leur environnement. En effet la nuit permettent à l'homme de s'extraire de sa vision anthropocentrique. De l'univers et de faire l'expérience du monde vivant non humain. Il est donc primordial de sauvegarder cet environnement nocturnes. Au niveau local, sa protection doit se faire de manière territorialisée en tenant compte des besoins, mais également des appréhensions, des concitoyens qui varie selon le sexe et les zones habitées, qu'elle soit justifiée ou non. Scientifiquement, plusieurs études ont montré qu'il y avait une réelle adhésion des concitoyens. Pour réduire l'intensité lumineuse et le nombre de points lumineux. Concrètement, il faut d'abord réfléchir à la finalité des éclairages et à leur réelle utilité et utiliser des technologies les moins impactante possible pour la diversité. À cet égard, les collectivités territoriales peuvent bénéficier depuis janvier 2023 et vous n'avez largement détaillé les aides du fonds Vert qui vise justement à concilier rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public et protection de la biodiversité, ainsi que réduction de la pollution lumineuse. Au-delà des pouvoirs publics, tous les acteurs privés participant à la pollution lumineuse doivent se mobiliser à travers une communication massive sur les règles à respecter et les bonnes pratiques en matière d'éclairage. Il s'agit des magasins de bricolage et de fabricants d'ampoules et de lampadaires qu'ils doivent informer et conseiller leurs clients dans le sens d'une optimisation de l'éclairage dans la durée et en quantité. Il s'agit des syndicats de l'éclairage ou encore des fédérations de commerçants qui doivent sensibiliser leurs adhérents sur la législation en vigueur. En conclusion je voudrais insister sur l'efficacité et la simplicité des mesures à prendre pour lutter contre la pollution lumineuse. Contrairement à d'autres pollutions comme la pollution chimique par exemple la pollution lumineuse et très facilement réversible. Il suffit d'éteindre la lumière pour protéger la biodiversité et nos écosystèmes sans oublier les économies d'énergie que cela génère, je nous encourage donc tous à prendre notre bâton de pèlerin et à sensibiliser les communes, les acteurs économiques et les citoyens pour protéger notre environnement nocturnes et garantir notre cohabitation avec le vent le monde vivant non humain. Je vous remercie pour votre attention. Merci cher collègue. Merci à tous les participants à ce débat. Merci madame la ministre. Mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance jeudi 13 avril, 2023 10h 30 pour les questions orales. La séance est levée.